sous les réserves d'usage. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue François Vendasi, qui fut sénateur de la Haute-Corse de 2005 à 2014. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (texte de la commission n° 137, rapport

en acceptant pour l'essentiel les ajustements, ouvertures et annulations de crédits proposés sur le budget de l'État, tout en notant que le déficit demeurait considérable, celui-ci se situant sur un « plateau » dont il paraissait bien difficile de redescendre. Le Sénat a également pris acte, sans s'opposer à la plupart d'entre elles, des mesures fiscales pérennes que l'Assemblée nationale a fait le choix d'adopter, revenant en cela sur une pratique établie depuis 2018, que nous retrouverons toutefois l'an prochain du fait de la révision de la loi organique relative aux lois de finances.

Autre dépense à noter, le soutien financier apporté à l'Ukraine, notamment sur la mission « Défense ». Nous y sommes bien entendu favorables. Les députés ont par ailleurs procédé utilement au doublement du seuil d'imputation du déficit foncier sur le revenu global pour les dépenses de rénovation énergétique,

Par ailleurs, la CMP a conservé le soutien à l'action des maisons France Services introduit par le Sénat pour permettre le développement et le bon fonctionnement de ces structures tout en limitant la charge pesant sur les petites collectivités,

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs,

budgétaires. Ce compromis trouvé entre l'Assemblée nationale et le Sénat est une bonne nouvelle pour les Français, confrontés chaque jour à la hausse des prix. Je veux saluer le travail mené

ce projet de loi de finances rectificative constitue une sorte de « rallonge », dans un contexte particulièrement difficile. Vous le savez, depuis le début de l'année, la vie chère met notre société à rude épreuve. Face à cette nouvelle donne, notre action peut se résumer en une phrase : tout faire- je dis bien tout faire -pour que la crise énergétique ne se transforme pas en une crise économique majeure. Pour cela, nous faisons un choix clair, celui de protéger les Français sans jamais accepter la dérive de nos comptes. Dépenser sans limites aujourd'hui signifierait moins de liberté d'action pour demain.

S'agissant de 2023, je veux partager avec vous une prévision encourageante publiée lundi par le Fonds monétaire international (FMI). L'institution table sur une croissance de 0,75 % pour notre pays, une prévision très proche de celle qui a été retenue pour construire le projet de loi de finances, qui marque la capacité de résistance de notre économie.

Concrètement, ce texte va permettre d'aider 12 millions de ménages qui se chauffent au gaz, à l'électricité, au bois ou au fioul à payer leurs factures. Nous mettons 1,8 milliard d'euros sur la table pour financer le chèque énergie exceptionnel, concrètement un versement de 100 ou de 200 euros qui sera effectué d'ici à la fin de l'année. J'en profite pour rappeler que la première LFR pour 2022 a déjà prévu un budget de 230 millions pour aider les ménages qui se chauffent au fioul. Cette aide commence à être déployée et se traduit par l'attribution d'un chèque de 200 euros pour les ménages déjà bénéficiaires du chèque énergie, et de 100 euros pour ceux des troisième à cinquième déciles.

Vous le savez, la Première ministre avait annoncé une prolongation jusqu'à la mi-novembre de la ristourne de 30 centimes par litre de carburant pour tenir compte du blocage des raffineries et des difficultés d'approvisionnement dont ont pâti nos compatriotes. cette prolongation, qui représente un coût pour nos finances publiques de l'ordre de 440 millions d'euros pour deux semaines. Depuis la semaine dernière, cette remise à la pompe a été réduite à 10 centimes par litre, comme nous l'avions annoncé. Pour autant, 2023 ne sera pas synonyme d'un arrêt brutal du soutien apporté aux automobilistes. La réalité, c'est que nous devons continuer à soutenir les travailleurs qui ont besoin de leur voiture. Il s'agit en effet d'agir de manière plus ciblée, en concentrant l'argent public sur celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Nous avons donc prévu un fonds de 275 millions d'euros, qui pourra être immédiatement débloqué au bénéfice des opérateurs du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans la même logique, ce PLFR prévoit l'ouverture de crédits pour les frais de carburant exceptionnels du ministère des armées : 200 millions d'euros sont ainsi débloqués pour nos militaires en opérations extérieures. Parce que les prix des produits alimentaires connaissent une inflation particulièrement forte,

Au total, ce sont donc 2,5 milliards d'euros qui sont mis sur la table pour aider les Français et certains opérateurs de l'État à faire face au choc énergétique. Mais il ne s'agit pas seulement de parer à l'urgence. Ce texte procède aussi à un certain nombre d'ajustements de fin de gestion, avec le souci permanent de tenir les comptes publics. publics. Les ouvertures de crédits auxquelles nous procédons pour assurer de nouvelles dépenses, de l'ordre de 5 milliards d'euros, sont donc compensées par des annulations de crédits d'un montant identique. Autrement dit, nous vous présentons aujourd'hui un texte d'équilibre budgétaire, hors dépenses exceptionnelles liées à la crise de l'énergie.

Autre ouverture significative : 1,1 milliard d'euros sont débloqués pour la mission « Défense » afin de financer le soutien militaire que nous apportons à l'Ukraine. Je souligne aussi les 100 millions d'euros supplémentaires issus d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale Charles de Courson, du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT), et Benjamin Haddad, du groupe Renaissance. Permettez-moi enfin de revenir sur les modifications introduites par le Sénat et retenues dans le cadre des travaux de la CMP. Je sais qu'il s'agit de sujets majeurs pour celles et ceux qui les ont portés, et plus largement pour l'ensemble de la Haute Assemblée. Nous avons intégré l'amendement qui prévoit d'abroger la réforme de la répartition du produit de la taxe d'aménagement entre les communes et leurs groupements. Je rappelle que l'article 109 de la loi de finances pour 2022

Nous avons choisi également d'accorder des moyens supplémentaires au financement de nos infrastructures, comme l'a souhaité le rapporteur général Jean-François Husson, avec 50 millions d'euros pour la rénovation des ponts

Tout cela, nous le finançons sans céder un pouce de terrain au laisser-aller budgétaire. En effet, 2022 n'a pas seulement été l'année du combat contre la vie chère ; ce fut aussi l'année du combat pour des comptes bien tenus, avec un déficit stabilisé à 5 % du PIB. Nous tenons

Cette maîtrise des comptes est possible grâce à une économie qui résiste, à l'engagement et au travail de chacun. Avec ce projet de loi de finances rectificative, nous aidons les Français à se chauffer et à se déplacer, nous aidons nos étudiants et nos chercheurs à travailler dans de bonnes conditions, nous soutenons les banques alimentaires, nous finançons la bataille en faveur du plein emploi et nous assumons notre choix de nous tenir aux côtés du peuple ukrainien.

sans recours au 49.3. Dans la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, sans majorité absolue pour la majorité présidentielle, ce n'était pas gagné d'avance

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

pour la rénovation ou la construction de ponts, la commission ayant notamment été inspirée par le travail de mon collègue Michel Dagbert, coauteur avec Patrick Chaize d'un rapport publié en 2019 sur la sécurité des ponts. Je salue de même les 100 millions d'euros supplémentaires débloqués pour accélérer la rénovation des réseaux d'eau et la réduction des fuites. salue également l'abrogation de la réforme de la répartition de la taxe d'aménagement entre les communes et leurs groupements, pour revenir à une situation plus simple, celle de la liberté des communes.

Je salue surtout l'augmentation de la part de l'État dans le financement des maisons France Services, pour atteindre l'objectif de 50 000 euros par établissement d'ici à 2023, à 2023, comme le proposait notre collègue Bernard Delcros dans son rapport. France Services est une réussite, qui porte ses fruits. Vecteurs de cohésion sociale, les services publics reviennent dans de nombreux territoires éloignés des métropoles. Nous atteindrons l'objectif de 2 500 maisons maisons France Services, avec un maillage de l'ensemble du territoire. L'attente est forte chez nos concitoyens, et je ne peux que me réjouir de cet effort qui s'inscrit dans le projet du Président de la République et du Gouvernement, à l'image des réouvertures de six sous-préfectures annoncées en octobre dernier. Comme je l'indiquais en première lecture, ce PLFR démontre ainsi que, lorsqu'un dialogue apaisé et constructif s'installe, le Parlement peut travailler sereinement sur un texte budgétaire et l'adopter, même en l'absence de majorité absolue, avec des amendements issus des oppositions. Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, l'a souligné lui-même : le texte final conserve « tous les amendements » que son groupe proposait, à savoir les aides pour les chaudières à bois, pour l'aide alimentaire et pour les communes qui souhaitent revaloriser les revenus de leur personnel soignant. Voter ce PLFR, c'est aussi voter les mesures historiques présentées par le Gouvernement pour faire face à la hausse des prix de l'énergie : le chèque énergie exceptionnel, qui concernera 12 millions de foyers, avec 200 ou 100 euros à la clef pour les ménages les plus modestes. bien sûr, la prolongation de la remise carburant de 30 centimes jusqu'au 15 novembre, pour un coût de 440 millions d'euros, puis de 10 centimes jusqu'au 31 décembre. Sur l'année 2022, cette aide sur le prix du litre de carburant représente au total 8 milliards d'euros, soit 30 millions d'euros par jour. Voter ce PLFR, c'est aussi voter le fonds de 275 millions d'euros pour aider les universités, les centres de recherche et les Crous, ou encore les 200 millions d'euros supplémentaires pour les achats de carburant des armées pour les opérations extérieures. Au total, ce budget rectificatif prévoit 2,5 milliards d'euros d'aides exceptionnelles pour faire face à la hausse des prix de l'énergie.

Je me félicite qu'un accord ait été trouvé entre les deux chambres. Alors que les 49.3 s'enchaînent, il est important de constater que, sur ce texte, la représentation parlementaire s'en sort par le haut.

En effet, auparavant, les communes pouvaient reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d'aménagement aux structures intercommunales. L'article 109 de la loi de finances pour 2022 est venu modifier les mots « peut-être » pour les remplacer par le mot « est ». Ce faisant, le reversement, jusque-là simple faculté pour les communes, est devenu obligatoire. Cette obligation de reversement niait le fondement même de la dynamique de coopération intercommunale. C'est à la commune de garder la capacité d'apprécier librement, en bonne intelligence avec l'intercommunalité, la pertinence d'un partage éventuel de la taxe d'aménagement avec l'EPCI, en fonction des équipements publics intercommunaux qu'elle accueille sur son territoire. Faire de cette faculté une obligation relevait de l'infantilisation des maires, à qui il fallait imposer ce que la loi leur permettait déjà de faire s'ils jugeaient une telle répartition légitime. Le nouveau texte vise à revenir à la situation antérieure à celle qui a été créée par l'article 109 de la loi de finances pour 2022 ; c'est louable.

Sur ce point, une étude du cabinet d'audit S&P estime que les collectivités locales vont perdre 3 milliards d'euros par an de budget avec la stabilisation de la dotation globale de fonctionnement (DGF), la suppression de la taxe d'habitation issue de la réforme de la fiscalité locale en 2021 et la suppression de la Monsieur le ministre, vous prévoyez que les collectivités locales contribuent pour un quart à la réduction des dépenses publiques de 2023 à 2027. Je le dis sans ambages, c'est pour elles un lourd fardeau, étant donné qu'elles ne représentent que 19 % des dépenses, 8 % de la dette et qu'elles n'ont pas de déficit. Je pense aussi que cela pourrait affecter négativement le tissu économique local, car il n'est pas inutile de rappeler que les collectivités représentent plus de 60 % de l'investissement public total. De fait, leur investissement devrait baisser de 12 % hors inflation d'ici à 2024 par rapport à son pic de 2019. Tous vos dogmes mènent donc à la baisse des impôts de production, qui, sous couvert de garantie de compétitivité des entreprises, n'ont de cesse de baisser. Car le mythe d'une spirale des petits entrepreneurs écrasés par la fiscalité locale n'existe pas. Cette baisse des impôts de production est en réalité la poursuite d'une logique plus générale de baisse des prélèvements, qui conduit à sacrifier l'investissement public sur l'autel de la compétitivité. Pour s'en convaincre, la littérature scientifique ne met pas en évidence un lien entre niveau de fiscalité et dynamisme des entreprises, et l'on sait que la création d'emplois par les entreprises dépend autant de leur lieu d'implantation, qui est modelé par l'investissement public, que de leurs caractéristiques individuelles. Vous le savez, la baisse des impôts de production affecte le financement de nos collectivités locales. Si l'État déclare la compenser à l'euro près, il devient malgré tout décideur et revient sur l'autonomie financière des collectivités. C'est précisément pour cette raison que, dans sa note, le Conseil d'analyse économique recommande d'affecter aux régions une part des recettes de la TVA en fonction du poids des collectivités dans la valeur ajoutée globale des entreprises. ce PLFR de fin de gestion va dans le bon sens. Néanmoins, parce qu'il traduit encore l'idéologie qui est la vôtre,

sémillant VRP de la politique gouvernementale. C'est votre rôle. La commission mixte paritaire a trouvé un accord sur le projet de loi de finances rectificative pour 2022. Chacun verra des avancées dans un texte dont la portée est toute relative. Il intègre des mesures qui arrivent trop tard, bien trop tard, ces retards étant la conséquence de choix inadaptés

très loin du compte. Autant d'angles morts qui n'ont pas vocation à figurer dans un projet de loi de finances rectificative : la rectification doit intervenir au moment de la loi de finances initiale, dont nous sommes en train de débattre, au pire par la voie d'un collectif budgétaire. À trop tarder,

Il y a, par ailleurs, ceux qui ont pu bénéficier des mesures du paquet pouvoir d'achat. Dans ce « paquet pouvoir de survie » adopté à l'été, les avancées étaient notoirement insuffisantes, on le constate aujourd'hui. Tant et si bien que le ministre se félicitait de « cette première étape », renchérissant en ces termes : « Le Gouvernement souhaite que nous puissions continuer dans cette voie au service de nos compatriotes. » Mais l'inflation se confirme, insistante- nous l'avons expliqué en première lecture -, et le Gouvernement s'est arrêté en chemin.

de l'année et qu'il se borne à un chèque énergie exceptionnel pour les ménages bien au-dessous des revenus médians. Nous répétons que la politique des chèques relève du saupoudrage, mais que, faute de mieux, nous les prenons. Il s'agit, je l'ai dit, de la survie de nombre de nos compatriotes. En ce qui concerne les collectivités territoriales, le collectif budgétaire revient sur la ponction, votée à l'Assemblée nationale, des recettes d'Ifer des départements. La logique en matière de fiscalité énergétique ne peut pas être celle des vases communicants, avec des transferts de l'un vers l'autre à périmètre constant. Les réformes de la fiscalité intervenues lors du précédent quinquennat ont complètement bouleversé l'équilibre et la cohérence des recettes des collectivités locales. Il n'est pas acceptable que la répartition du produit des recettes fiscales ait pour conséquence, dans notre République, la mise en concurrence des différents échelons territoriaux. Il faut penser Il faut penser leur complémentarité et refondre une fiscalité au plus près des compétences. Sans cela, la lutte fera rage pour déterminer qui devra récupérer le produit de l'autre. Ce sera un combat sans fin, au détriment de l'action publique territoriale si nécessaire.

Des mesures importantes ont été adoptées pour permettre aux Français de passer la période hivernale plus sereinement, compte tenu du contexte inflationniste que nous subissons tous. Je n'y reviendrai pas dans le détail, mais je pense au versement des chèques énergie pour les ménages les plus précaires

Les motifs de satisfaction du groupe Union Centriste sont nombreux. Outre les mesures que je viens d'aborder, nous nous félicitons que cette CMP conclusive ait pu retenir des dispositions significatives adoptées par le Sénat.

Le financement des maisons France Services a été forfaitisé- on le sait -à hauteur de 30 000 euros par an. Or le coût moyen de fonctionnement d'une maison France Services est d'environ 110 000 euros. Pour répondre à cette situation, notre collègue Bernard Delcros a fait adopter

de délibérer sur l'affectation d'une fraction du produit de la taxe d'aménagement à leur EPCI. Ce dispositif contrariait, me semble-t-il, le fondement même de la dynamique de coopération intercommunale. Enfin, je veux souligner l'ouverture de 20 millions d'euros de crédits afin de financer les projets d'insonorisation destinés aux riverains des aéroports et, ainsi, de lutter contre les nuisances sonores aéroportuaires. Alors que le rendement de la taxe sur les nuisances sonores aériennes a connu une très forte diminution depuis 2020 en raison de la baisse du trafic sur laquelle elle est assise, la perte de financement cumulée pour ce dispositif pouvait s'élever à plus de 80 millions d'euros l'année prochaine. C'est pourquoi le déblocage de 20 millions d'euros que j'ai proposé est un signal

par la voix de son rapporteur général, que je remercie au passage pour la qualité et le sérieux de son travail. En 2019, notre collègue centriste Hervé Maurey avait présidé une commission d'enquête sur sur la sécurité des ponts et appelé à un véritable plan Marshall en faveur des ponts du bloc communal. On sait que les ponts routiers des collectivités territoriales sont dans un état parfois préoccupant, notamment dans les plus petites communes, qui, bien souvent, n'ont pas les moyens de les entretenir.

Le texte enrichi par le Sénat et les sénateurs centristes ayant été largement intégré dans la version issue de la CMP qui nous est présentée, le groupe Union Centriste adoptera ce PLFR à la quasi-unanimité.

comme cap la bonne gestion de nos finances publiques. Si ces mesures se conçoivent aisément au vu de l'urgence de la situation, elles n'en demeurent pas moins coûteuses. Aussi, je rappelle que nous devons nous attaquer au redressement rapide de nos finances publiques,

sur le second projet de loi de finances rectificative pour 2022, qui s'équilibre sans recours à l'emprunt, ce qui est rare et mérite d'être souligné.

Mais permettez-moi d'entrer directement dans le vif du sujet en évoquant les points qui constituent de réelles avancées pour les collectivités territoriales. Tout d'abord, la décision de revenir sur la réforme de la taxe d'aménagement au bénéfice des EPCI me paraît satisfaisante,

Cette mesure aligne l'Ifer photovoltaïque sur l'éolien et contribue à davantage de cohérence et de clarté, même si j'aurais souhaité une part plus importante pour les communes.

du réseau routier, la CMP en a retenu 50. Quant aux 100 millions de subventions exceptionnelles votées par le Sénat pour les agences de l'eau afin de contribuer à réduire le taux de fuite et à rénover les réseaux d'eau, la CMP n'en retient que 50 millions.

ce qui représente environ 5 000 euros par structure et permet de maintenir un partage des charges à 50 % entre l'État et les collectivités locales. Nous devons être vigilants, car, trop souvent par le passé, le partage du financement entre État et collectivités locales a été oublié.

Comme toujours, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Pour ma part, je retiens de l'examen du texte issu de la CMP sur le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2022 le rôle central du Sénat, reconnu comme partenaire des collectivités territoriales. En responsabilité et tout en gardant en tête le nécessaire cap du redressement des comptes publics, ce dernier a en effet permis de donner au bloc communal les moyens de faire face à ses missions en cette période très difficile.

de fin de gestion de la part du Gouvernement, il a également été amendé et travaillé avec sérieux par les deux chambres de notre Parlement. Il contient donc, faut-il le noter, des avancées significatives pour les Français et les collectivités territoriales. le Sénat a réussi à s'accorder avec l'Assemblée nationale sur un texte qui comporte notamment une enveloppe de 2,5 milliards d'euros d'aides supplémentaires pour faire face à l'inflation et à la crise énergétique. égard, je le redis : une réponse européenne est attendue sur les prix, la réponse budgétaire ne pouvant être durable. La sagesse de notre Haute Assemblée ne s'est pas arrêtée à la confirmation des annonces gouvernementales. Nous avons aussi proposé de nouvelles dispositions en faveur de nos territoires. Ainsi, nous avons débloqué 50 millions d'euros pour la réfection des ponts et du réseau routier, dont les besoins sont aujourd'hui très importants pour des raisons de sécurité et de bonne circulation. Si vous

Nous avons également voté l'accélération de la rénovation des réseaux d'eau, par une subvention exceptionnelle accordée aux agences de l'eau à hauteur de 50 millions d'euros. les sécheresses de l'été 2022 ont endommagé les infrastructures du réseau d'eau déjà fortement abîmées, puisqu'on estime que, chaque année, 20 % du volume d'eau potable distribuée chez les usagers est perdu, ce qui représente un milliard de mètres cubes d'eau. cubes d'eau. Sur l'initiative de la commission des finances, nous avons aussi voté l'augmentation de 12,5 millions d'euros des crédits dédiés au financement des maisons France Services. Cela permettra d'assurer un appui renforcé à leur fonctionnement, pour que ces guichets de proximité, qui regroupent plusieurs administrations, soient des lieux d'accompagnement de nos concitoyens dans tous les territoires et soient, à terme, financés à hauteur de 50 000 euros par maison. Enfin nous avons ajouté une nouvelle dotation destinée aux travaux d'insonorisation des riverains des grands aéroports à hauteur de 20 millions d'euros. Je me félicite par ailleurs que l'amendement que j'ai eu l'honneur de porter ait été voté et retenu par la CMP. Il permet de rétablir la situation prévalant avant 2022 quant à l'affectation du produit de la taxe d'aménagement au sein du bloc communal au seul bénéfice de la commune, dans le respect des libertés locales et des pactes financiers territoriaux qui peuvent ensuite se nouer.

les aspects techniques de l'abrogation et nous confirmer notamment que les délibérations déjà prises cette année seront bien automatiquement abrogées. Je tiens également à souligner les apports de nos collègues du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui ont défendu notamment la prorogation en 2023 de l'attribution de MaPrimeRénov'sans

pour notre pays, pour peu que le Gouvernement entende et accepte les propositions qui lui sont faites. Avant de conclure, je tiens à remercier au nom de mon groupe le travail de notre rapporteur général, qui a permis d'aboutir à cet accord. Nous savons le rythme de travail auquel il est soumis lors du marathon budgétaire de fin d'année. Mes remerciements vous sont également adressés, monsieur le ministre, pour l'écoute dont vous faites preuve. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera ce second projet de loi de finances rectificative pour 2022, tel qu'il ressort des conclusions de la CMP. La parole

je me réjouis à mon tour que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord sur le deuxième projet de loi de finances rectificative de l'année. C'est un coup double pour l'année 2022 : après l'adoption du paquet pouvoir d'achat cet été, l'Assemblée nationale et le Sénat sont de nouveau parvenus à élaborer un texte commun au bénéfice des Français. Permettez-moi, néanmoins, de commencer par une brève remarque critique, qui rejoint les propos du rapporteur général. Par sa voix, la commission des finances du Sénat a regretté que le véhicule du PLFR de fin d'année que nous examinons en même temps que le PLF pour l'année 2023 intègre des mesures fiscales nouvelles, notamment pour 2023, contrairement à la vocation première d'un PLFR. le Gouvernement avait fait preuve d'une rigueur appréciable, en vidant les collectifs budgétaires de fin d'exercice des mesures budgétaires et fiscales les plus lourdes. Cela permettait de concentrer les débats de PLFR sur les ajustements classiques et nécessaires en fin d'exercice. Cette méthode a le mérite de clarifier les choses, j'espère que nous pourrons bientôt l'appliquer de nouveau. Je ne reviendrai pas sur les grands équilibres de ce texte, qui n'ont pas évolué de manière significative au cours des débats. Nous sommes parvenus à maintenir le déficit public à 5 % du PIB, malgré des dépenses supplémentaires votées par les deux chambres, et ce grâce à des recettes plus dynamiques que prévu, ce qui confirme la résilience de notre économie. Ces recettes supplémentaires ont notamment permis de financer le chèque énergie exceptionnel. Cette aide, d'un montant de 100 à 200 euros, concerne les ménages les plus modestes. Bien sûr, la politique du chèque a des défauts et des limites que je ne m'attarderai pas à rappeler- bon nombre de nos collègues s'en sont déjà chargés. Je tiens toutefois à saluer le fait que ce chèque soit ciblé sur les plus modestes, même si le ciblage demeure assez large, puisque 40 % des foyers y sont éligibles. Le ciblage des mesures de soutien au pouvoir d'achat matérialise le passage du « quoi qu'il en coûte » au « combien ça coûte ». Les certitudes sur le présent et, surtout, les incertitudes sur le futur nous obligent à aborder les dépenses publiques avec davantage de prudence. Je n'ai pas pour habitude de me réjouir des dépenses publiques supplémentaires, mais il est une ouverture de crédits prévue par ce projet de loi de finances rectificative que je tiens à saluer. Il s'agit du renforcement de l'aide militaire de la France à l'Ukraine. Ces crédits supplémentaires font suite aux engagements pris par le Président de la République. Au total, ce texte apporte 1,1 milliard d'euros pour financer l'aide que nous apportons aux hérauts de la liberté que sont les Ukrainiens. Il est indispensable que la France poursuive son soutien matériel à l'Ukraine, car un soutien moral sans soutien matériel, c'est un peu comme un chèque en bois : à la fin, on perd en crédit bien davantage que ce qu'on espérait gagner. Ce qui se joue à l'Est est bien davantage que la paix en Europe, ce qui est déjà immense ; c'est la survie de la démocratie face aux dictatures. Il ne faut pas faiblir. Je me réjouis que personne, notamment à l'Assemblée nationale, n'ait appliqué à ces crédits une lecture strictement comptable. Cela aurait soit révélé une courte vue, soit dénoncé de coupables accointances. Une grande partie de nos dépenses publiques nouvelles, et donc des sacrifices que les Français consentent, soit aujourd'hui par l'inflation, soit demain par l'impôt, sont indirectement le fait du boucher du Kremlin, ne l'oublions pas.

Le chèque énergie exceptionnel ou encore l'aide exceptionnelle aux ménages se chauffant aux pellets ou à la bûche sont également de bonnes mesures, parce qu'elles sont des mesures ciblées en direction des ménages les plus modestes, et c'est essentiel. Nous saluons aussi les différentes avancées obtenues en commission mixte paritaire, comme l'augmentation du budget consacré à l'aide alimentaire ou encore la possibilité, pour les communes, de revaloriser les revenus du personnel soignant. Certains apports du Sénat ont été maintenus, bien que revus à la baisse, comme les crédits nécessaires débloqués pour la réfection des ponts et du réseau routier ou la subvention exceptionnelle accordée aux agences de l'eau, qui est tout aussi nécessaire. cette liste non exhaustive montre que, quand le Gouvernement écoute, quand vous laissez le temps au dialogue parlementaire, nous pouvons arriver à des compromis. D'ailleurs, le compromis serait encore meilleur si vous écoutiez plus de l'oreille gauche. Cependant, Cependant, en miroir à l'examen du PLF dont nous venons de terminer la discussion de la première partie, nous déplorons toujours que l'écologie ne soit pas le coeur des projets et des budgets. Nous vous avons proposé quelques mesures écologiques et sociales, comme l'exonération de TVA sur l'usage domestique des premiers mètres cubes d'eau, soit la quantité jugée vitale par J'entends bien que toucher à la TVA est contraire au droit européen, mais, chers collègues, l'accès à l'eau pour les besoins élémentaires est un droit fondamental. Il faudra donc changer les choses pour que les besoins de base ou le fait de remplir sa piscine Le plafonnement de la hausse des prix de l'énergie à 15 % prévu par le bouclier tarifaire a des effets positifs, mais demeure d'une faible efficacité en matière de justice écologique et sociale. C'est le sens de la demande de rapport que nous avons faite sur une tarification duale, qui protégerait davantage les ménages en deçà d'un seuil de consommation et les soumettrait au prix de marché au-delà. Nous vous avons également proposé de soutenir les collectivités par l'amortissement de la revalorisation du point d'indice sur trois ans. Vous avez balayé cette proposition d'un revers de main. Je veux donner deux exemples concrets. À Grenoble, cette revalorisation conduit à une hausse de la masse salariale de 2,7 millions d'euros en 2022 et de 5 millions en année pleine. À Arcueil, la hausse Les collectivités savent gérer de nouvelles charges, mais, lorsqu'on leur impose une trajectoire sur cinq ans inférieure à l'inflation, l'exercice devient périlleux,

Je terminerai mon propos sur ce PLFR, texte technique de fin de gestion, en vous invitant de nouveau à vous pencher sur la question de la résilience de notre pays et sur la nécessité de penser chaque mesure d'urgence du point de vue de la résilience. Les mesures de court terme peuvent être nécessaires. Elles peuvent panser des plaies et stopper des hémorragies, mais elles ne suffisent pas. Notre planète est malade, malade de notre suractivité, de notre surconsommation et de notre surcompétitivité, qui consiste parfois à créer des produits en France, les fabriquer en Chine et les ramener par bateau dans notre pays. Il est urgent de changer de modèle.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'examen du budget de la mission « Sécurités » pour 2023 s'inscrit dans un contexte qui pourrait appeler à la nouveauté d'une part, il s'agit du premier budget du second quinquennat du président Emmanuel Macron ; d'autre part, c'est également le premier budget de mise en oeuvre des annonces faites dans le cadre du projet de loi d'orientation et de Pourtant, en examinant précisément le budget de la mission, on constate avant tout une forme de continuité. Certes, il y a des changements positifs qu'il faut souligner. Globalement, les crédits de la mission sont ainsi en hausse et je m'en réjouis. de Lopmi prévoit d'ailleurs une hausse cumulée du budget du ministère de l'intérieur de 15 milliards d'euros entre 2023 et 2027. En 2023, pour ce qui concerne l'ensemble de la mission « Sécurités », la hausse des crédits s'élève à 1,43 milliard d'euros en crédits de paiement, soit une hausse d'un peu moins de 7 %. Pour la police et la gendarmerie nationales, les crédits de paiement sont en hausse de 1,34 milliard

En 2023, ces crédits sont en particulier dédiés à la modernisation numérique et à l'équipement de la gendarmerie et de la police nationales. C'est une dynamique nécessaire. S'agissant du numérique, il est notamment prévu, d'une part, de développer les outils numériques des forces de sécurité intérieure afin d'améliorer leurs conditions de travail et favoriser leur présence et leur efficacité sur le terrain, de renforcer les moyens de lutte contre la cybercriminalité, en augmentant par exemple le nombre de « cyberpatrouilleurs », et d'améliorer la relation numérique avec les citoyens. Par ailleurs, l'équipement des policiers et gendarmes fait également l'objet d'efforts pour assurer l'opérationnalité de nos forces et accompagner les hausses d'effectifs. Est notamment prévu en 2023 le renouvellement des équipements de protection, d'intervention et de maintien de l'ordre, de l'habillement et des outils technologiques de pointe. La tenue de la Coupe du monde de rugby en 2023 et la préparation des jeux Olympiques de 2024 justifient cet effort sur l'équipement de nos forces. Pour autant, comme je le disais, le présent budget présente aussi des caractéristiques de continuité ; on pourrait même dire qu'il retombe dans certains travers constatés par le passé, ce que l'on peut regretter. En premier lieu, on constate une stabilisation de la part des dépenses de personnel dans l'ensemble des dépenses de la police et de la gendarmerie en 2023. C'est une mauvaise nouvelle, d'autant qu'une dynamique de baisse avait été amorcée en 2021. Comme je l'ai souvent rappelé, il est indispensable de réduire la part des dépenses de personnel dans l'ensemble du budget des deux forces, afin de dégager des marges de manoeuvre suffisantes pour l'équipement et l'investissement. Or il est souvent arrivé dans le passé que les dépenses de personnel dérapent au détriment de l'investissement et des autres dépenses de fonctionnement. En 2023, 83 % des autorisations d'engagement et 86 % des crédits de paiement seront consacrés aux dépenses de personnel pour les deux forces- c'est beaucoup. Cette stabilisation de la part des dépenses de personnel s'explique par le fait que ces dernières augmentent de 5,8 % pour les deux forces en 2023. Cette hausse provient, d'abord, de la poursuite de la politique de recrutement. Comme vous le savez, le Président de la République a décidé la création de plus de 10 000 emplois de 2018 à 2022. Alors que ce plan de création de postes était achevé, la Première ministre, Élisabeth Borne, a annoncé, le 6 septembre la création de 8 500 postes de policiers et de gendarmes d'ici à 2027, poursuivant ainsi sur la lancée du quinquennat précédent. Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit la création de 2 857 pour les deux forces, dont 1 907 pour la police nationale et 950 pour la gendarmerie nationale. Ces recrutements ont nécessairement des conséquences financières notables. En outre, l'année 2023 sera également marquée par le coût lié à la revalorisation du point d'indice de la fonction publique intervenue au 1 juillet 2022, pour un coût d'environ 170 millions d'euros pour les deux forces. Enfin, le poids des mesures catégorielles atteindra, en 2023, 85 millions d'euros pour la police nationale et 72 millions pour la gendarmerie nationale. Ce montant est en forte hausse du fait des premières conséquences budgétaires des deux protocoles conclus en mars 2022. et c'est la deuxième limite du présent budget, les crédits de la mission sont insatisfaisants s'agissant de certaines dépenses de fonctionnement et d'investissement. Le risque est, comme cela est déjà arrivé par le passé, qu'à la sortie d'un plan d'équipement porté cette fois-ci par le plan de relance les dépenses d'investissement se tarissent, dans une sorte de difficilement soutenable. En particulier, l'investissement dans l'immobilier ne répond pas à l'acuité des enjeux, surtout pour la gendarmerie nationale. En effet, les crédits d'investissement portés par la mission pour les locaux de la gendarmerie, c'est-à-dire principalement les casernes, sont en baisse de 42,5 millions d'euros en autorisations d'engagement. Ils n'augmentent que très modérément, de 13,5 millions d'euros, en crédits de paiement. Globalement, les crédits de paiement s'établissent ainsi à 130 millions d'euros

Le caractère modeste de cette somme doit être souligné, d'autant qu'à compter de 2023 les crédits du plan de relance ne viennent plus apporter un complément significatif comme cela avait été le cas en 2021 et 2022. Je rappelle que, s'agissant de l'immobilier, l'effort doit être maintenu sur la durée.

3 219 personnes ayant alors été tuées sur les routes de France. Par rapport à 2019, cependant, année de référence avant la pandémie, la mortalité avait diminué de 9 % et l'accidentalité, de 4,5 %. Le bilan sur les sept premiers mois de 2022 présente quant à lui une augmentation de la mortalité routière par rapport à 2019. Les recettes et les crédits du CAS sont en hausse de 7 %.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaiterais, en préambule de mon intervention, rendre hommage à l'ensemble des sapeurs-pompiers, des pilotes et des formations militaires de la sécurité civile et des associations agréées tous s'investissent sans compter dans la lutte contre les crises qui touchent notre pays, comme nous l'avons de nouveau constaté cet été, marqué par des feux de forêt d'une ampleur quasi inégalée. Ces incendies ont rappelé à quel point notre modèle de sécurité civile doit être préservé. Je me félicite à cet égard de la hausse importante des crédits du budget du programme 161 pour l'année 2023.

qui permettront, dans le cadre de cofinancements entre l'État et les collectivités locales, de soutenir des projets d'investissement au bénéfice des Sdis. Un montant de 30 millions d'euros sur cinq ans devait initialement leur être consacré, ce qui apparaissait particulièrement faible au regard des besoins d'investissement des Sdis. Le Gouvernement a toutefois procédé à un renforcement bienvenu de cette dotation durant l'examen de ce PLF, en l'abondant d'un montant de 150 millions d'euros, dont 37,5 millions au titre de l'année 2023. Le Président de la République a néanmoins indiqué, lors de ses annonces du 28 octobre dernier, que cette dotation de 150 millions d'euros s'inscrivait dans le cadre de la compensation de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. On ne peut donc pas présenter cette enveloppe comme un véritable renouvellement de l'effort de l'État en faveur du financement des Sdis, puisqu'elle consiste en réalité en une réaffectation aux Sdis d'une recette qui bénéficiait déjà à leurs principaux financeurs, à savoir les collectivités locales. Malgré cette réserve, on ne peut que se féliciter de la concrétisation de ces pactes capacitaires dans un contexte où les Sdis doivent investir massivement pour se doter des moyens de faire face à l'augmentation des sollicitations opérationnelles. J'en viens maintenant à la question du nécessaire renforcement de la flotte aérienne de la sécurité civile. Ce projet de loi de finances pour 2023 contient plusieurs avancées à cet égard. Je me félicite tout d'abord du renouvellement et de l'extension à venir de notre flotte d'hélicoptères Dragon vieillissante et amputée ces dernières années de plusieurs appareils à la suite d'accidents tragiques.

Ces hélicoptères, contrairement à ceux de la flotte actuelle, seront équipés d'une capacité de largage d'eau importante et pourront dès lors être utilement mobilisés pour la lutte contre les feux de forêt. Le vieillissement de la flotte de canadairs constitue également une source de préoccupation partagée depuis plusieurs années par l'ensemble des acteurs de la sécurité civile. Les annonces faites par le Président de la République le 28 octobre dernier d'un renouvellement intégral et d'une extension de cette flotte se sont traduites par un amendement du Gouvernement visant à financer une commande d'une douzaine d'appareils. Cette commande est évidemment bienvenue, mais le calendrier de livraison des canadairs suscite des interrogations : la chaîne de production de ces avions, à l'arrêt depuis plusieurs années, vient à peine d'être relancée et les premiers appareils ne pourront probablement pas être livrés avant 2027. Il est donc important que le ministère de l'intérieur identifie d'autres pistes de renforcement de la flotte à court terme. Il me semble par ailleurs que l'enjeu du renforcement des moyens aériens de la sécurité civile ne peut être envisagé sous le seul prisme capacitaire. Les problématiques de prévention des feux de forêt, du dimensionnement des infrastructures d'accueil des aéronefs ou de la disponibilité des moyens humains nécessaires au fonctionnement opérationnel de la flotte doivent également être prises en considération. Or la direction générale de la sécurité civile est confrontée à de grandes difficultés pour recruter et fidéliser ses pilotes d'aéronefs. Cette profession souffre indéniablement d'un déficit d'attractivité en moyenne, un pilote de la sécurité civile est trois fois moins payé qu'un pilote de l'aviation commerciale. Le présent PLF prévoit certes des mesures de revalorisation pour les personnels navigants, estimées à 1,5 million d'euros, mais je souhaiterais vous entendre, madame la ministre, sur la stratégie envisagée par le ministère de l'intérieur pour pallier ces difficultés de recrutement et renforcer l'attractivité de la profession de pilote de la sécurité civile. Je conclurai mon propos en évoquant le projet de mutualisation des systèmes d'information des Sdis : NexSIS 18-112. Les nombreux retards dans le déploiement du projet ont conduit à entamer la confiance des Sdis dans sa concrétisation. Cette situation fragilise le modèle économique de NexSIS, puisque les Sdis sont largement impliqués dans le financement du programme par l'intermédiaire de leurs contributions volontaires. Ces contributions devraient être complétées par un soutien renforcé de l'État en faveur de l'Agence du numérique de la sécurité civile, dont les moyens sont aujourd'hui bien trop faibles pour permettre le déploiement du projet dans de bonnes conditions. En tout état de cause, les investissements consentis dans le cadre de ce budget pour 2023 vont indéniablement dans le bon sens. Pour cette raison, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter les crédits de la mission « Sécurités ». La parole

pour avis. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après plusieurs années de progression des crédits de la gendarmerie nationale due notamment au plan de relance, nous pouvions craindre un retour de balancier. Grâce à la programmation prévue dans le cadre du projet de Lopmi, ce n'est pas le cas. Nous pouvons donc saluer des des crédits globalement en hausse en 2023 : ils passent de 9,3 milliards à 9,9 milliards d'euros en crédits de paiement, soit une hausse de 6,4 %. En outre, les effectifs progresseront de 950 emplois, permettant la création de 7 escadrons de gendarmerie mobile et le début de la mise en place de 200 nouvelles brigades territoriales. Celles-ci seront sans doute regardées comme un apport très utile dans certains départements après des années de suppression et de regroupement de brigades. Il est vrai que, lors de l'examen du projet de Lopmi, nous avions exprimé quelques interrogations à ce sujet.

préoccupation sur la capacité des collectivités territoriales à investir pour construire des locaux. Outre les dispositifs de soutien existants au travers des décrets de 1993 et de 2016, la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) a été évoquée. Madame la Madame la ministre, avez-vous prévu des dispositifs supplémentaires, conformément à l'amendement adopté par le Sénat au sein du rapport annexé au projet de Lopmi ? D'autres aspects de ce budget représentent à notre sens un progrès indéniable, en particulier les 120 millions d'euros de crédits de paiement pour la modernisation informatique et la création d'une agence du numérique des forces de sécurité intérieure. Je rappelle qu'en 2019 nous avions eu des interrogations sur la création d'une direction du numérique

Pouvez-vous nous confirmer, madame la ministre, que la nouvelle agence du numérique sera bien construite à partir du STSI, mais avec davantage de moyens ? Pour le reste, le budget du programme 152 pour 2023 affiche une certaine stagnation des crédits hors titre 2 après plusieurs années d'efforts dans ce domaine. S'agissant de l'investissement immobilier, la Lopmi a prévu la mise en place d'un nouveau service chargé de planifier les nouvelles constructions et la maintenance lourde selon un échéancier qui reste à élaborer. que nous serons très attentifs à cette question. En conclusion, le budget de la gendarmerie nationale pour 2023 affiche une nouvelle progression des crédits, permettant de poursuivre la mise à niveau numérique, la montée en puissance des effectifs et une présence accrue auprès des populations.

qui permettront de poursuivre la modernisation de la gendarmerie, en mettant en oeuvre les nouvelles étapes de NÉO et du système PC Storm, qui constitue une brique essentielle du réseau Radio du futur. Tous ces nouveaux systèmes numériques génèrent logiquement des dépenses récurrentes pour le maintien en condition opérationnelle et le renouvellement des équipements. Cela montre une fois de plus l'importance de la programmation pluriannuelle. difficile de tout financer à la fois, mais il ne faut pas laisser se dégrader un aspect pendant que l'on en renforce un autre. Développer les meilleurs outils numériques, c'est bien, mais si parallèlement les gendarmes exercent dans des brigades décrépites et sont logés dans des casernes dégradées, c'est problématique et inacceptable. ne prévoit pas de programmation des investissements permettant de remédier à ces points noirs bien connus. Une fois de plus, les investissements prévus pour l'immobilier au sein du programme 152 seront insuffisants en 2023. Avec un montant de 126 millions d'euros, on est loin des 300 millions annuels nécessaires. L'année dernière, un effort avait pourtant été accompli pour passer de 100 millions d'euros à 150 millions- on revient donc en arrière. Le Sénat a pourtant adopté notre amendement au sein du rapport annexé au projet de Lopmi, prévoyant ce nécessaire investissement de 300 millions d'euros annuels dans l'immobilier domanial. Quelle est votre intention, madame la ministre, s'agissant de la mise en oeuvre de cette disposition, pour 2023 mais aussi pour les années suivantes ? En ce qui concerne les véhicules, un renouvellement de 2 000 unités seulement est prévu pour 2023, chiffre le plus bas depuis 2014. qu'un effort important avait été consenti sur la période 2020-2022, avec plus de 3 500 véhicules par an, ce qui a permis de rajeunir un peu le parc.

nous serons bien au-dessous du renouvellement annuel de 10 % du parc pourtant inscrit dans le rapport annexé au projet de Lopmi. Je terminerai par un point positif, en évoquant la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Le projet de Lopmi prévoit le passage de 30 000 à 50 000 réservistes, objectif qui paraissait ambitieux compte tenu de la stagnation des crédits au cours des dernières années. Or on observe bien, au sein du programme 152 pour 2023, une hausse de 20 % des crédits fléchés vers la réserve, ce dont nous nous félicitons. La progression significative des crédits du programme 152 a conduit notre commission à donner un avis favorable sur leur adoption, même si nous gardons à l'esprit certains points négatifs, en particulier la poursuite du sous-investissement dans l'immobilier auquel il faudra impérativement remédier dans les prochaines années.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission des lois a donné un avis favorable sur l'adoption des crédits de la mission « Sécurités ». Ce projet de loi de finances fait suite à plusieurs années de larges concertations-

Ce projet porte des ambitions programmatiques fortes pour le budget du ministère de l'intérieur, puisque ce ne sont pas moins de 15 milliards d'euros supplémentaires qui seraient budgétés sur cinq ans par rapport aux crédits affectés au ministère Tant les dépenses de personnel que de fonctionnement et d'investissement augmentent en 2023, ce qui permettra de financer les priorités fixées par le projet de Lopmi. La commission a toutefois assorti de trois réserves son avis favorable sur l'adoption des crédits. La première concerne la prise en compte de l'inflation de Lopmi a été élaboré avant la survenue de ce phénomène et les budgets n'ont pas été revalorisés en conséquence. La police et la gendarmerie nationales vont donc devoir participer à l'effort national de rationalisation des dépenses, mais cela ne devra pas porter préjudice à la capacité des forces à faire face aux échéances de 2023 et 2024. Deuxième réserve, le doublement des effectifs sur la voie publique n'aura de sens que si les effectifs des services judiciaires qui traitent les enquêtes et ceux des juridictions sont augmentés de manière proportionnelle. Sans cela, c'est toute la chaîne pénale qui serait engorgée sans amélioration de la réponse pénale. Enfin, Enfin, la troisième réserve concerne la nécessaire diminution de la part des dépenses de personnel dans le budget global de ces deux programmes : après deux années de diminution nette, cette tendance est moins claire en 2023. Une évolution structurelle est nécessaire

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission des lois a donné un avis favorable sur l'adoption des crédits du programme 161 relatif aux moyens nationaux de la sécurité civile. Nous saluons la hausse significative tant des autorisations d'engagement, qui dépassent pour la première fois le milliard d'euros, que des crédits de paiement. Ces crédits supplémentaires permettront de renouveler et de renforcer notre flotte d'hélicoptères, conformément aux préconisations formulées l'année dernière par la commission des lois. Cette forte hausse nous paraît nécessaire, et même vitale, tant l'année 2022 a mis à rude épreuve tous les acteurs de la sécurité civile. Avec 72 000 hectares brûlés, soit sept fois plus que la moyenne annuelle des vingt dernières années, la dernière saison des feux a marqué une nette rupture dans notre appréhension des aléas, remettant en question de nombreuses certitudes quant à la résilience de notre modèle de lutte contre les incendies. de manière urgente. Outre la réquisition précipitée de huit hélicoptères, la France, qui traditionnellement aide ses voisins, a eu recours, pour la première fois depuis son instauration en 2001, au mécanisme européen de protection civile. Nous avons donc incontestablement atteint les limites capacitaires de nos forces de sécurité civile. C'est pourquoi notre avis favorable ne s'apparente aucunement à un quitus à l'égard du Gouvernement. Tout d'abord, nous insistons sur la forte attente de notre part quant à la publication, par le Gouvernement, du rapport sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, demandé dans le cadre de la loi visant En effet, toute réflexion générale sur les moyens de la sécurité civile, rendue nécessaire cette année, doit impérativement associer les collectivités territoriales et se pencher sur l'enjeu du financement des Sdis, mis en difficulté par l'ampleur de la dernière saison des feux et ne disposant pas des mêmes leviers financiers que l'État pour y répondre. Absolument ! Concernant les moyens aériens nationaux, nous avons émis de vives réserves quant aux effets d'annonce autour du plan de renouvellement et de renforcement des canadairs, largement commenté par le ministre de l'intérieur à l'occasion de l'examen puis décrit comme une nouveauté lors du discours du Président de la République le 28 octobre dernier. Cela fait en outre plus de trois ans que sont attendus les deux canadairs devant être commandés dans le cadre de l'Union européenne et pourtant mis en avant dans tous les discours gouvernementaux sur la sécurité civile. Par ailleurs, le calendrier ambitieux, affiché par le Président de la République, visant un renouvellement intégral de nos canadairs d'ici à la fin du quinquennat paraît irréaliste, alors qu'aucun financement n'a encore été engagé. Cela démontre une certaine confusion dans la communication gouvernementale à deux reprises, le ministre de l'intérieur a déclaré à notre commission qu'il y avait de fortes tensions sur la chaîne de production des canadairs et que ceux-ci devront se faire attendre plusieurs années, même en faisant preuve d'optimisme. Nous serons donc particulièrement vigilants

une mise à niveau des équipements : acquisition de gilets tactiques, développement de solutions opérationnelles comme le PC Storm, pour permettre aux forces de sécurité de communiquer un outil unique et sécurisé,

n'a de sens que si les effectifs des services judiciaires traitant les enquêtes et des juridictions sont augmentés proportionnellement. Il y a un lien direct, chacun le comprend bien.

Marc. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le budget que nous examinons aujourd'hui reprend les éléments du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, voté en lecture il y a peu. Ce texte prévoit une augmentation des moyens consacrés à nos forces de l'ordre. La progression de l'insécurité doit en effet être enrayée. C'est le souhait non seulement du Président de la République, mais aussi, je le crois, de tous les citoyens de ce pays. Il s'agit bien sûr d'accroître la présence policière sur le terrain,

Il sera cependant nécessaire d'envisager une réforme en profondeur de la procédure pénale, afin de la simplifier. Tous les acteurs du monde judiciaire en bénéficieront, les justiciables au premier chef. Pour accroître cette présence, il faut aussi augmenter les effectifs. C'est notamment ce que permettent les crédits de la mission « Sécurités ». Entre 2017 et 2022, plus de 8 000 policiers et plus de 2 000 gendarmes ont été recrutés, 10 000 agents supplémentaires qui veillent à la sécurité de nos concitoyens et de nos entreprises, ainsi qu'à la sûreté de nos territoires. Cette dynamique se poursuit cette année encore, et nous nous en félicitons. Ainsi, près de 3 000 emplois seront créés en 2023. En plus d'une augmentation d'effectifs, nos forces de l'ordre ont besoin d'investissements massifs, en matière tant d'équipement que d'immobilier. Les policiers et les gendarmes exercent un métier dangereux, dans des conditions difficiles et tendues. Aussi, ils doivent pouvoir compter sur un matériel de qualité. La question du parc automobile est un sujet sensible, même si l'on peut constater, ces dernières années, que la situation

Les délits de fuite sont de plus en plus nombreux et entraînent de plus en plus de dégâts. Les policiers et les gendarmes doivent être en mesure de maîtriser les suspects. Ils ont pour cela besoin de véhicules puissants, fiables et, donc, récents. au renouvellement de la flotte de véhicules. Le parc immobilier a, lui aussi, grand besoin d'être rénové et modernisé. La dynamique est enclenchée. Il convient de maintenir cet effort dans la durée. Les missions des forces de l'ordre évoluent sans cesse. À mesure que le numérique prend une place de plus en plus importante dans nos vies, la délinquance et le crime s'y développent. Nos policiers et gendarmes doivent acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles capacités pour faire face et assurer la sécurité de nos concitoyens. Nous avons tous en tête les récentes attaques informatiques qui ont ciblé des hôpitaux ou encore des communes. La complexité et l'impact de ces opérations ne cessent de croître. Parallèlement, de récentes arrestations ont mis au jour d'importants réseaux pédopornographiques dans notre pays. Tout cela révèle l'ampleur prise par le numérique dans le travail des forces de l'ordre. Le projet de Lopmi prévoit, en conséquence, un plan de modernisation numérique, particulièrement nécessaire et attendu. Au-delà de ces nouveaux champs d'intervention, policiers et gendarmes assurent également des missions plus classiques, mais tout aussi importantes. J'évoquerai plus particulièrement la sécurité routière. Ce sujet ne fait pas les gros titres des journaux, mais les accidents de voiture emportent chaque année la vie de plus de 3 000 de nos concitoyens, c'est-à-dire trois fois plus que le nombre d'homicides. L'augmentation des crédits dédiés à la sécurité routière est donc bienvenue, d'autant que 2022 semble être une année particulièrement mauvaise à cet égard. Il faut inverser la tendance.

première traduction financière du projet de Lopmi, présenté par ce gouvernement, le budget de la mission « Sécurités » voit les crédits alloués à ce volet de l'action publique fortement augmenter. Nous devrions nous en réjouir, mais nous ne sommes pas là pour ne regarder que le chiffre en bas du tableau. C'est bien la répartition et l'utilisation de ces fonds qui interrogent notre groupe. Lors des longs débats que nous avons eus autour du projet de loi de programmation, nous avons pu exposer notre vision des forces de l'ordre : au service des citoyens et au plus proche d'eux. Lors de cet examen, nous avons bien voté l'article comprenant la trajectoire d'augmentation des crédits alloués aux serviteurs de l'État,

Ce sentiment d'abandon, de manque de moyens, d'accompagnement, de formation, aggravé par la politique du chiffre et des missions aussi chronophages qu'inutiles, se traduit, hélas, par l'épuisement de nos forces de l'ordre. 24 % des gendarmes ou policiers déclarent être confrontés à des pensées suicidaires. C'est cela qui devrait être la priorité. Nous avons bien perçu la continuité d'une politique, plus répressive que protectrice, qui ignore tant les liens de confiance à renforcer avec la population que que cette immense souffrance au travail de nos forces de l'ordre, lesquelles s'engagent pourtant pour agir auprès de la population, avec la population, pour la population. Ce gouvernement préfère allouer l'argent public à la numérisation, à une robotisation outrancière, une modernisation de façade, qui oublie les problèmes du quotidien, à la fois des citoyens et des agents. et des agents. La numérisation ne simplifie la vie que d'une partie de la population : l'illectronisme est une réalité qui touche 13 millions de personnes en France. Ne les laissons pas à la porte de nos services publics

nous nous réjouissons du renforcement des services de lutte contre la cybercriminalité. Nous saluons l'ensemble des agents qui ont récemment permis l'interpellation de plusieurs cyberpédocriminels.

un développement de façade d'une police structurée autour du tout-répressif ; une multiplication de nouvelles compagnies de CRS calibrées, nous dit-on, pour faire face aux grands événements que notre pays s'apprête à accueillir, mais sans repenser notre doctrine de maintien de l'ordre, qui a pourtant brillé par sa médiocrité devant le monde entier lors d'un grand événement L'évolution des dépenses de fonctionnement et d'investissement entre la police et la gendarmerie diffère : elles augmentent ainsi significativement pour la police nationale, mais diminuent pour la gendarmerie nationale. Nous défendons une police de proximité, essentielle pour renouer le lien de confiance avec les citoyens. Ce sont donc bien les missions que l'on doit questionner avant l'allocation des moyens. Le tout-répressif et la culture du chiffre ont leurs limites, mais ce budget est loin de dresser un tel constat. Pour ce qui est des missions inutilement consommatrices de forces et de moyens, l'exemple de la lutte contre le cannabis est emblématique de l'impasse d'une politique antidrogue inefficace. Malgré tous les coups de filet, les points de démontés, toutes les amendes forfaitaires, vous vous heurtez toujours au même problème : les Français aiment ce produit et en sont toujours parmi les plus grands consommateurs d'Europe. Votre politique ne tient que par votre dogmatisme et ne fait qu'épuiser les troupes.

Sur le volet sécurité civile, notre déception est grande. Comme partout ailleurs, les moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux liés au changement climatique. Ils ne permettent pas de construire une première ligne solide face aux périls qui viennent. Le budget de la sécurité civile n'est de nature, selon nous, ni à répondre au besoin réel de prévenir les risques accrus à venir ni à compenser les dégâts subis cet été. Le renforcement des moyens de lutte contre les incendies est bienvenu, certes, mais son niveau est insuffisant dans un contexte inflationniste. Dans l'ensemble, ce budget ne nous convient pas. Nous restons dubitatifs, au même titre que le Conseil d'État, qui a également déploré un manque de données sur la situation et l'évolution des phénomènes d'insécurité et de délinquance au cours des dernières années, ainsi qu'une absence d'évaluation des dernières lois sécuritaires adoptées depuis 2018. Aussi, notre groupe ne pourra voter les crédits de la mission « Sécurités ».

que, dans les commissariats ou services de sécurité publique des grandes agglomérations, nous manquons d'encadrants stables. La gestion des carrières est un levier efficace

bénie -où il y avait un accord de fond entre les collectivités, principalement les départements, et la gendarmerie nationale, pour assurer le financement en capital des installations et la récupération de ces investissements sous s'est dégradé, parce que le prix des installations de gendarmerie a crû très substantiellement dans les années qui ont suivi. Aujourd'hui, l'équation financière ne fonctionne plus. Il me semble que c'est un petit défi pour le ministère de travailler à une standardisation et à une homogénéisation des plans des locaux de gendarmerie, de sorte que les collectivités investisseuses

qu'une première compagnie de location de trottinettes avait décidé de le faire de sa propre initiative. Cela signifie que l'État a laissé passer un train.

conformément à la trajectoire contenue dans le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, qui a animé nos débats voilà quelques semaines. Dont acte ! Si l'on peut se féliciter

crédits alloués à la sécurité et à la paix publiques, à la sécurité routière ainsi qu'aux missions de police judiciaire et concours à la justice subissent tous des baisses de plus de 13 %.

Trois audits commandés par M. Darmanin et M. le garde des sceaux n'ont pas encore livré leurs résultats. Ces travaux devraient, je l'espère, être utiles pour rassurer la police judiciaire partout sur le territoire national.

notre vote ne signifie pas une adhésion sans réserve. Nous avons par ailleurs entendu les voix qui nous disaient que seule la rationalisation budgétaire avait guidé cette réforme. Nous serons donc vigilants, chaque année, à la bonne application de la prochaine Lopmi, qui donne des moyens supplémentaires à nos forces de sécurité, mais nous nous attacherons également à ce que la réforme de la police judiciaire ne conduise pas à de nouvelles difficultés de résolution des affaires. C'est une question de respect des droits de nos concitoyens. En ce qui concerne la gendarmerie, le projet de loi de programmation sanctuarise la dynamique ascendante de ses crédits. Tant mieux ! Le renforcement des moyens de la police et de la gendarmerie se traduit par la poursuite des recrutements

Ce recrutement doit pouvoir garnir les rangs des nouvelles brigades rurales et des nouveaux escadrons de gendarmerie mobile qui ont été annoncés. Notre groupe soutient bien évidemment ces mises en place et va même plus loin : nous porterons ainsi un amendement à allouer 50 millions d'euros supplémentaires aux gendarmeries rurales, et ce afin d'anticiper une révision du décret de 1993 sur les subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie. Rappelons-le, aux termes du projet de Lopmi, la police et la gendarmerie doivent doubler leur présence sur la voie publique, notamment en vue de la Coupe du monde de rugby en 2023 en 2023 et des jeux Olympiques en 2024. L'intégration de nouvelles recrues va mettre en tension les capacités de formation, d'autant que s'y ajoute l'intégration de la formation d'officier de police judiciaire au cursus des gardiens de la paix, toujours aux termes de ce même projet de loi.

n'assure donc qu'une part minoritaire du financement du budget total des Sdis. Cela dit, pour 2023, la participation de l'État augmente de 13 %, dans le droit fil des objectifs contenus dans le projet

les grands défis auxquels les pompiers doivent faire face du fait du dérèglement climatique nous imposent de leur accorder des moyens à la hauteur de leur mission. Quant

négative. Nous demandons qu'il appartienne au législateur d'apprécier au cas par cas et dans le respect de ce principe la pertinence du recours à cette procédure, au regard de la conciliation à opérer entre la nature du délit concerné, la protection des droits des personnes mises en cause et des victimes, la défense des intérêts de la société et les exigences tant d'une bonne administration de la justice que d'une répression effective des infractions. Voilà ce qui doit conduire notre parcours législatif.

moi l'idée de diaboliser la dématérialisation ou de sous-estimer sinon sa nécessité, du moins son utilité pour accéder à des informations et effectuer des démarches administratives, mais elle ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la relation entre

ne doit pas se faire au prix d'une rupture du lien entre citoyens et police. De plus, les crédits de l'action Missions de police judiciaire et concours à la justice, qui regroupe l'ensemble des activités de police judiciaire et des missions

Nous déduisons de son manque d'envergure que la départementalisation de la police nationale aura de lourdes conséquences sur la police judiciaire. Dénoncée tant par les professionnels de la sécurité que par ceux de la justice,

et à la création du Centre national de formation cyber (CNF-Cyber), qui assurera la formation continue des enquêteurs spécialisés- c'est évidemment indispensable.

du Sénat, la réforme engagée en 2011 de la défense extérieure contre l'incendie (DECI) « n'a pas tenu ses promesses et a provoqué un large mécontentement de la part des maires : 70 % des maires interrogés par la Délégation estiment que la concertation n'a pas été suffisante et du département de l'Orne

». Cette multiplication des inquiétudes et des dangers résonne bien avec le pluriel employé dans l'intitulé de cette mission, dont les enjeux sont singulièrement variés. En premier lieu, il y a la sécurité quotidienne : celle de la vie ordinaire de nos concitoyens, des rues et des lieux publics,

à l'approche de deux événements phares : la Coupe du monde de rugby et les jeux Olympiques. En troisième lieu, il y a la sécurité de crise : je pense en particulier aux incendies de cet été, qui ont durement frappé la Gironde. Durant ces moments, les agents doivent être mobilisés sans discontinuer.

saluons l'affectation de crédits supplémentaires en vue de développer les outils de lutte contre les cybercriminalités. Il ne faut nullement négliger cette question. Le piratage au cours de l'été du réseau informatique de l'hôpital de Corbeil-Essonnes a montré avec force la nécessité de poursuivre l'investissement dans ce domaine. enfin : je ne peux que saluer les crédits qui devraient être alloués au renouvellement de la flotte d'hélicoptères. Nous voyons donc que, afin d'assurer toutes ces missions de sécurité publique, il nous faut des agents et du matériel en nombre suffisant.

Je le redis : qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation continue, trop souvent délaissée au cours de la carrière, il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la performance des différents services.

amendements visant à encourager l'investissement dans la lutte contre l'incendie. Je pense notamment à la proposition de notre collègue Jean-Yves Roux d'accompagner financièrement les communes rurales dans la réalisation de leurs obligations légales de débroussaillement, encore à l'amendement de Nathalie Delattre visant à financer l'acquisition de drones, utiles à la lutte contre les incendies. Ces remarques faites, notre groupe devrait voter en faveur des crédits alloués à cette mission.

est essentielle pour tous les Français. Elle détermine les moyens mis à la disposition de l'État pour assurer l'une de ses missions premières : garantir à chacun de nos concitoyens le droit à mener une vie tranquille dans notre pays, à y vivre en sécurité. dans mon propos, mesdames, messieurs les sénateurs, quelques réponses aux questions que vous avez soulevées. Beaucoup a été fait depuis 2017, sous la conduite du Président de la République, pour renforcer la sécurité intérieure. Des efforts budgétaires constants ont été consentis, se traduisant, par exemple, par le plan de recrutement exceptionnel de 10 000 policiers et gendarmes, ou encore

dans le cadre, notamment, du Beauvau de la Sécurité, qui s'est achevé au mois d'octobre dernier. Ce projet de loi d'orientation et de programmation prévoit une hausse du budget du ministère de 15 milliards d'euros sur cinq ans. Cette augmentation historique n'est pas seulement l'addition de moyens nouveaux ; elle est mise au service d'une vision stratégique refondée de la sécurité intérieure, portée par le PLF pour 2023.

Au travers de la mission « Sécurités », nous nous donnons les ressources nécessaires pour intensifier et améliorer encore les constantes de l'action publique : notre lutte contre la criminalité et toutes les formes de délinquances, la prévention des risques et la prise en charge de nos concitoyens en danger. Cela passe par le renforcement de nos capacités opérationnelles et par l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des agents de la sécurité intérieure. Nous nous donnons également les moyens d'apporter une réponse forte et adaptée aux défis inédits auxquels la France fait face en ce moment, dans un contexte de multiplication des crises à la fois géopolitiques, économiques, sociales, environnementales Autant de menaces nouvelles pour nos concitoyens, qui risquent, à terme, si nous n'en prenons pas la pleine mesure, de déstabiliser notre contrat social et de mettre en péril la cohésion de la Nation. La mission « Sécurités » comporte quatre programmes distincts, qui recouvrent les différents volets de l'action de l'État en matière de sécurité intérieure. Au total, comme dans chacune de ses parties, la mission « Sécurités » porte un engagement financier en nette augmentation par rapport à l'année dernière. budget global de la mission est en hausse de 6,82 % en autorisations d'engagement et de 6,65 % en crédits de paiement par rapport à 2022.

l'objectif premier est bien de répondre au besoin d'une présence accrue d'agents sur la voie publique, conformément à l'objectif fixé par le Président de la République d'en doubler le nombre en dix ans. Continuer à déployer davantage d'agents sur le terrain revient à améliorer directement la qualité de vie de nos concitoyens dans tous les territoires, en métropole comme en outre-mer.

de force mobile parisiennes qui seront libérées de leurs missions de garde statique. Ces nouveaux agents renforceront également les circonscriptions de sécurité publique prioritaires de la police nationale. Ils seront déployés en particulier sur la voie publique et dans les transports en commun.

En parallèle, nous accompagnerons la montée en puissance de la réserve opérationnelle de la police et de la gendarmerie nationales, l'objectif étant d'atteindre 50 000 réservistes d'ici à 2027. Le budget spécifiquement consacré à la réserve de la gendarmerie sera crédité de 14 millions d'euros, soit un renfort de 6 000 réservistes, tandis que celui de la réserve de la police sera abondé à hauteur de 8 millions d'euros.

Le PLF pour 2023 vise également à donner les moyens nécessaires au ministère de l'intérieur dans la perspective de la Coupe du monde de rugby et des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Pour les jeux Olympiques, le ministre vous a présenté, d'octobre, le détail du dispositif de sécurisation envisagé pour cet événement inédit : près de 35 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en moyenne par jour.

concomitant, est d'affermir l'ancrage territorial de nos forces de sécurité intérieures, afin de résorber les zones blanches sécuritaires qui peuvent exister dans notre pays.

Cette solution de télécommunication résiliente et interopérable est un atout indispensable pour permettre à nos forces de sécurité de gagner en efficacité.

Nous poursuivons également le déploiement de la vidéoprotection sur la voie publique, pas moins de 22 millions d'euros étant programmés à cet effet pour la seule année 2023.

est la prise en compte croissante des nouvelles frontières de la délinquance, en particulier numériques. La filière cyber sera ainsi renforcée grâce au recrutement de 1 500 gendarmes et policiers cyberpatrouilleurs supplémentaires et au développement d'un appel d'urgence, le « 17 cyber ». d'urgence, le « 17 cyber ». Ensuite, le déploiement dès l'année prochaine des premiers éléments de la gendarmerie verte, formée aux atteintes à l'environnement et dotée d'un commandement unique, L'année 2023 amorcera également la première étape de la mise en place des protocoles sociaux liés à la mise en oeuvre de la Lopmi, qui visent à améliorer de façon substantielle les conditions de travail de tous les agents de la sécurité intérieure. des mesures d'aide en matière de logement pour les policiers, mais également des aides à la garde d'enfants en horaires atypiques, les premières revalorisations de grilles indiciaires et l'augmentation de certaines primes et d'indemnités, comme la prime qui était attribuée aux officiers de police judiciaire, l'indemnité journalière d'absence temporaire ou encore la prime pour le travail de nuit des policiers. Premier acte de la Lopmi, cette mission « Sécurités » témoigne, vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, de notre volonté d'en engager résolument la dynamique, au service de nos forces de sécurité et d'une meilleure protection de nos concitoyens, en particulier à l'approche des grands rendez-vous sportifs et populaires que notre pays accueillera dans les prochains mois. Le même volontarisme se retrouve dans le programme « Sécurité civile ». Cette année, plus encore que les années précédentes, les conséquences du réchauffement climatique se sont cruellement fait sentir sur notre territoire. Je pense aux feux de forêt dévastateurs de cet été, aux ravages de la tempête Fiona en Guadeloupe ou encore aux fortes intempéries qu'ont connues la Somme et le Pas-de-Calais récemment. Face à ces menaces d'ampleur, nous devons réarmer notre sécurité civile pour lui permettre de faire face à des crises toujours plus complexes et inattendues dans les années à venir. Les objectifs déjà importants fixés dans la première version du programme 161 seront encore augmentés par deux amendements gouvernementaux, afin d'inclure les dernières mesures annoncées par le Président de la République en retour d'expérience de la saison de feux de forêt.

Les engagements pris dans le cadre de cette enveloppe exceptionnelle ouverte en 2023 donneront lieu à des paiements étalés au cours des prochaines années, au fil du déploiement des projets d'investissement mis en oeuvre par les collectivités territoriales au profit des Sdis.

Le nombre de tués sur les routes de France a continué de diminuer en 2021 par rapport à 2019, dernière année de référence sans restriction de circulation, cette diminution Pour pérenniser cet élan, il faut bien sûr continuer d'agir en matière de dépistage et de formation, et pour cela recruter des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière supplémentaires. Il faut surtout agir en matière de prévention et de communication auprès de nos concitoyens. C'est une nouvelle fois l'axe fort de ce programme, pour cette année 2023, qui prend en compte de manière croissante les nouveaux facteurs d'accidentalité comme les mobilités douces.

Comme l'écrivait Henri Fayol, « prévoir, c'est à la fois supputer l'avenir et le préparer ; prévoir, c'est déjà agir ». C'est ce que cette mission permet de faire. Mesdames, messieurs les sénateurs, c'est à vous désormais qu'il appartient de la voter, au nom de l'intérêt général de notre pays et de nos concitoyens.